Les moyens des collectivités concernent la vie quotidienne de chacun dans nos territoires. Aussi cette question revêt elle une importance particulière pour nous, au Sénat, chambre des territoires, pour les élus locaux engagés chaque jour sur le terrain au service de leurs concitoyens, mais aussi pour tous les Français, bien au delà de la situation des collectivités elles mêmes. s’inscrit non dans une posture corporatiste, mais bien dans une logique d’intérêt général et de justice territoriale. Il y va de nos services publics de proximité et du quotidien, mais aussi de l’investissement public et de l’emploi dans notre pays. Le niveau global des contributions des collectivités à l’effort de redressement des comptes publics s’élèverait pour 2025, au terme de nos débats, à 2,2 milliards d’euros, au lieu des 5 milliards d’euros initialement proposés par le Gouvernement.

surtout insister sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico), que nous proposons d’instaurer et que nous avons adopté ce matin en commission des finances. Il s’agit d’un dispositif de mise en réserve des moyens de la collectivité, une sorte d’épargne forcée dans un compte au Trésor, qui n’est donc pas confiscatoire et qui permet de réduire le volume global de la dépense publique, améliorant ainsi notre solde public. ainsi notre solde public. Ainsi, l’effort réel des collectivités sera ramené à 1,2 milliard d’euros, tandis que les mesures fiscales qui les concernent, sans parler des décisions sectorielles s’attachant aux départements, peuvent produire encore davantage.

sans jamais atteindre 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Très bien ! Les autres éléments de la mission s’inscrivent dans une grande stabilité, malgré le contexte. L’article 61 porte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2025, en particulier des composantes péréquatrices de cette dotation, à hauteur de 300 millions d’euros.

L’article 63 porte diverses mesures de répartition de la fiscalité afférente aux déchets radioactifs, un sujet important pour les territoires de la Meuse et de la Haute Marne, qui sont les premiers concernés.

nous proposons donc de le supprimer purement et simplement et de lui substituer un dispositif nouveau n’opérant aucun prélèvement de ressources au profit de l’État, mais visant uniquement à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales qui sont en mesure de contribuer au redressement des comptes publics.

et de ses agences, en particulier, et renforcement de la décentralisation comme de l’État territorial. Dans notre pays, la dépense des collectivités ne représente que 19 % de la dépense publique totale, contre 34 % en Europe. En conclusion, la commission des finances a donné un avis favorable sur l’adoption des crédits de la mission et du compte de concours financier, modifié par son amendement de crédit ; elle donne également un avis favorable sur l’adoption de l’article 61, sous réserve de l’adoption de son amendement, ainsi qu’à l’adoption des articles 62 et 63

le vœu que nous puissions poursuivre ce travail en l’approfondissant, en abordant la réforme de la commande publique et la construction d’un véritable contrat de confiance autour des libertés locales et de la capacité d’agir des élus locaux, en responsabilité, avec une visibilité renforcée, dans un respect réciproque et au service des Français.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Les collectivités ont toujours su assumer leurs responsabilités et méritent d’être considérées comme de véritables partenaires pour porter les politiques publiques, et non comme de simples variables d’ajustement budgétaire.

Je ne le crois pas. Si je tiens à saluer le travail mené par mon collègue Stéphane Sautarel, qui tente de rendre ce dispositif moins inacceptable, je ne puis pour autant y souscrire. C’est dommage ! Cette année, nous vous présenterons donc cette mission

pour 2025, quand les transferts de l’État sont estimés à près de 104 milliards d’euros et même à 151 milliards d’euros au sens large, si l’on inclut les fractions compensatrices de TVA accordées en contrepartie des réformes fiscales. Les crédits du programme 119, qui portent les dotations de soutien à l’investissement local, ainsi que les dotations de décentralisation, ont été maintenus en autorisations d’engagement à leur niveau de 2024 et enregistrent une légère hausse en crédits de paiement. Ainsi, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) et la dotation politique de la ville (DPV) restent stables par rapport à la loi de finances initiale pour 2024 il en va de même des dotations générales de décentralisation des communes, des départements et des régions. Enfin, le projet de loi de finances ne revient pas sur les hausses récentes de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales (DSCAR), qui ont vu chacune leurs crédits rehaussés à 100 millions d’euros. Pour mémoire, la DTS avait été augmentée par le projet de loi de fin de gestion pour 2023, afin de traiter l’afflux des demandes de titres d’identité dans un délai raisonnable, et son montant avait été repris en loi de finances initiale pour 2024.

et moi même souhaitons saluer une réforme qui s’inscrit dans le sens des conclusions du rapport d’information de la commission des finances sur le verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. territoriales. La DSCAR offre désormais une reconnaissance de l’importance du travail réalisé par les communes rurales dans les zones classées. Elle gagnerait sans doute à être étoffée, et la commission a voté en première partie un amendement pour en porter le niveau à 110 millions d’euros. Beaucoup d’entre nous partagent ce satisfecit, mais souhaitent augmenter le nombre de communes bénéficiaires ou en modifier les critères de répartition. Assurément, cette nouvelle dotation pourra être évaluée de manière à identifier de nouveaux axes d’amélioration.

aussi parce que ces crédits s’inscrivent dans un projet de loi de finances qui, dans son ensemble, demande un effort sans précédent aux collectivités pour combler un déficit que celles ci n’ont pas créé.

devront, en effet, faire face dans les prochaines années à des investissements colossaux, d’une part, pour leurs bâtiments, afin de répondre aux enjeux du réchauffement climatique et de la transition écologique, et, d’autre part, dans les transports, pour répondre aux nécessités de nouvelles mobilités.

Cette loi, issue de la mission d’information du Sénat sur le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique, permet désormais de diminuer de moitié le reste à charge de la collectivité maître d’ouvrage et, ainsi, de mieux mobiliser les fonds alloués par l’État. Je souhaite enfin aborder l’avancée du plan Marseille en grand, notamment son volet concernant l’école, pour lequel une dotation dédiée de 250 millions d’euros avait été ouverte en loi de finances initiale pour 2022, au sein du programme 119. Dans le cadre de notre mission d’information réalisée cette année sur le sujet, nous avions émis des doutes sur la capacité de la Société publique des écoles marseillaises, créée dans le cadre dudit plan, à engager les consultations, lancer les travaux et livrer les équipements dans un délai prévu entre 2025 et 2031. de sa montée en charge se confirme, puisque, avec 56,8 millions d’euros inscrits en crédits de paiement au PLF pour 2025, l’ensemble des paiements effectués depuis 2022 atteindra 125 millions d’euros, soit moins de la moitié de l’enveloppe de 250 millions d’euros que j’ai mentionnée. Les raisons ayant poussé au lancement de ce plan restent néanmoins plus que jamais d’actualité, et j’appelle les élus à faire le nécessaire pour que celui ci puisse être mené à son terme. Enfin, les crédits du programme 122, qui concernent essentiellement les aides destinées à soutenir les collectivités faisant face à des situations exceptionnelles, enregistrent simultanément une forte baisse. Cette évolution résulte essentiellement de l’extinction des autorisations d’engagement pour le fonds de soutien exceptionnel pour les collectivités touchées par la tempête Ciaran.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, dans le cadre de ce marathon budgétaire, nous sommes appelés à examiner la mission « Relations avec les collectivités territoriales

le montant des crédits de cette mission reste faible. Toutefois, cette relative stabilité ne doit pas occulter le contexte général des finances locales, et particulièrement la participation au redressement des comptes publics qui est demandée aux collectivités locales. Je tiens à rappeler la position de la commission des lois à cet égard : si nos collectivités doivent effectivement prendre part à l’effort budgétaire, leur mise à contribution doit être juste et proportionnée. C’est pourquoi je défendrai, au nom de la commission des lois, un amendement tendant à supprimer le fonds de réserve prévu à l’article 64. Par cohérence et en responsabilité,

Ce dispositif est plus acceptable que le mécanisme prévu initialement : il ne prévoit aucun prélèvement de ressources au profit de l’État, mais vise uniquement à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales qui sont en mesure de contribuer au redressement des comptes publics, au travers d’une prise en compte plus fine de leur capacité contributive.

Pour finir, je profite du temps qui me reste pour interpeller le Gouvernement sur la question des dotations de soutien aux collectivités victimes de catastrophes naturelles. Indéniablement, une réforme en profondeur est indispensable au regard des limites du système actuel, qui conduit le Gouvernement, à chaque aléa climatique, à déployer en urgence en urgence des crédits exceptionnels pour venir en soutien des collectivités concernées. La ministre Françoise Gatel a ainsi annoncé jeudi dernier une enveloppe de 48 millions d’euros en faveur de quatre départements sinistrés, dont celui des Hautes Alpes, que je représente à la Haute Assemblée.

d’un homme qui, le soir des élections européennes, a décidé seul de dissoudre l’Assemblée nationale ; d’un homme qui, pendant tout l’été, a choisi, seul, de reporter de plus de

Ce jeu de l’opposition systématique entre les petits et les grands, entre les ruraux, les urbains et les périurbains, entre les territoires métropolitains et ultramarins, fracture et divise chaque jour un peu plus la République.

tous vos élus vous le disent : le compte n’y est pas, loin de là, et le Gouvernement y a contribué avec l’aide du parti Les Républicains, avec l’aide de votre majorité et, bien entendu, en cherchant à faire des concessions au Rassemblement national. Certes, les départements ont été un peu entendus,

nous dressons également le constat d’une raréfaction et d’une complexification des ressources fiscales et financières, faisant des finances locales un système imprévisible, illisible et inaccessible pour les élus des plus petites collectivités, d’autant que ces derniers n’ont aucune vision prospective à moyen terme des sommes qui leur seront allouées.

ci porte un budget jugé injuste par les Françaises et Français. Non ! Ce gouvernement n’a pas su écouter nos propositions responsables, parmi lesquelles

et aujourd’hui politique, ce projet de loi de finances prendrait la mesure de l’urgence de la responsabilité qui incombe à l’État. Ce n’est, hélas ! nullement le cas. Cette mission budgétaire s’inscrit dans une autre logique, celle d’un affaiblissement continu de l’autonomie et des moyens des collectivités, qui sont pourtant les premiers amortisseurs sociaux. C’est une logique centralisatrice, par laquelle l’intelligence locale est souvent sacrifiée.

témoigne, hélas ! d’un accord sur le fond. Cette année encore, il est demandé aux collectivités de faire toujours plus avec toujours moins. Nous ne pouvons que regretter cette contradiction flagrante entre les discours décentralisateurs et les actes centralisateurs de l’exécutif. Pour rappel, les crédits de cette mission représentent seulement 8 % des concours financiers de l’État aux collectivités et 4 % du total des transferts financiers. Ils ne recouvrent donc qu’une faible partie des crédits alloués aux collectivités locales.

cette stabilité est toutefois conditionnée à un verdissement croissant des dotations que nul ici ne conteste et que mon groupe soutient. Le Gouvernement a décidé d’attribuer jusqu’à 35 % de certains crédits à des projets liés à la transition environnementale.

faisons confiance à nos élus locaux, qui sont pragmatiques et responsables, pour définir leurs priorités. Leur imposer ce cadre rigide, c’est méconnaître leur capacité d’initiative et de discernement.

En tant qu’élu régional, je ne puis qu’attester le rôle primordial que jouent les régions dans l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, le développement économique, alors que leur budget est continuellement pressurisé. décembre 2023 de finances pour 2024, les dotations des régions ont diminué de 467 millions d’euros, soit près d’un tiers de leur montant. Comment continuer à parler de décentration lorsque les régions ne peuvent plus remplir leurs missions ? ils subissent aujourd’hui un effet ciseaux préoccupant. Leurs recettes stagnent, voire régressent, tandis que leurs dépenses sociales explosent. En 2023, plus d’un tiers d’entre eux ont vu leur épargne brute chuter fortement, réduisant d’autant leurs capacités d’investissement.

aux articles rattachés. L’article 64 portant création du fameux fonds de réserve illustre parfaitement les écueils de cette mission. Ce mécanisme, qui prévoit de prélever jusqu’à 3 milliards d’euros sur les recettes fiscales des grandes collectivités, repose sur des bases arbitraires et injustes. Non seulement il ne tient pas compte des situations financières spécifiques, mais il s’appuie sur des données passées, alors que les budgets ont été votés sans anticiper ce prélèvement.

en soit des négociations sur ce dispositif, nous ne pouvons pas souscrire à ce rabais qui concourt à l’asphyxie des collectivités territoriales.

mes chers collègues, à l’heure où l’État demande aux collectivités de contribuer à hauteur de plus de 8 milliards d’euros

de la République, dite loi NOTRe, la décentralisation est un bateau sans boussole. Les grandes régions n’ont pas apporté les économies attendues, et encore moins la proximité et l’efficacité de l’action publique locale ; les départements, dont d’aucuns projetaient la suppression, sont aujourd’hui pris à la gorge par des actions sociales obligatoires au périmètre élargi, avec des ressources sans cesse plus réduites les communes, enfin, sont intégrées de force dans des intercommunalités technocratiques, dépossédant les maires de leur pouvoir réel et abandonnant les citoyens dans des schémas et des actions incompréhensibles. Par ailleurs, le système de financement des collectivités a été désintégré. La suppression de la taxe d’habitation, mesure électoraliste présentée de manière illusoire comme un geste social fort, a distendu le lien entre le contribuable local et ses élus. Le transfert d’une part sans cesse croissante de la TVA aux régions et aux départements place ces collectivités sous le joug de l’État, les faisant passer d’un état d’autonomie pourtant reconnu constitutionnellement à un état de dépendance dans les faits. Chacun attend les futures élections municipales avec inquiétude. Combien de maires ne souhaiteront pas se représenter ? Comment les quelques citoyens dévoués parviendront ils à compléter les listes ? Et comment les futurs édiles, reconduits ou nouveaux,

et créent un fossé sans cesse plus grand entre les citoyens et les collectivités locales, qui constituent pourtant la première ligne de notre démocratie. La proposition par laquelle Gouvernement entend mettre à contribution les collectivités locales dans le cadre de l’effort de redressement des comptes publics n’est pas acceptable en l’état.

nous conduit à nous pencher sur les financements accordés par l’État aux collectivités locales. Les différents crédits de cette mission visent à soutenir l’investissement local et à permettre aux collectivités d’assurer les nouvelles compétences transmises dans le cadre de la politique de décentralisation. Ils regroupent également les subventions destinées à soutenir ponctuellement les collectivités confrontées à des circonstances exceptionnelles. La stabilité des crédits de cette mission

Les communes, qui réalisent 70 % des investissements publics de notre pays, sont le moteur de cette dynamique. Ces investissements concernent tous les domaines : écoles, équipements sportifs, infrastructures de transport, projets culturels ou encore actions environnementales. Ils participent directement du dynamisme économique local, en mobilisant les entreprises, en créant des emplois et en stimulant l’innovation. La dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales voit ses crédits pour 2025 maintenus au même niveau qu’en 2024, ce qui est une bonne chose. Ces crédits, destinés aux communes rurales dont une grande partie du territoire est composé ou situé à proximité directe d’une aire marine protégée et qui supportent ces charges de ruralité, leur permettent de jouer un rôle essentiel dans la protection de l’environnement et le développement durable de leur territoire.

Ces événements tragiques pour les territoires concernés montrent l’importance d’un accompagnement rapide et adapté. Je salue le courage et la résilience des élus locaux, en particulier des maires, qui se trouvent en première ligne face à ces crises

collègues. Compte tenu des très fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur notre pays, le groupe Les Indépendants – République et Territoires estime toutefois urgent de réduire les dépenses de l’État. S’il ne faut pas priver les collectivités de leurs capacités d’investissement, elles doivent que l’État et l’ensemble de ses organismes, en modérant leurs dépenses et en mettant en place des mécanismes permettant de faire face aux difficultés prochaines. L’article 64 du PLF prévoit ainsi la création d’un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales. ci sera alimenté par des prélèvements effectués auprès des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal excèdent 40 millions d’euros. Ces collectivités contribueraient à hauteur de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, indépendamment de leurs capacités contributives. Ce fonds permettra d’abonder, pendant les trois années suivantes, trois fonds de péréquation. Si nous soutenons un effort partagé et indispensable, ce mécanisme doit être soutenable et l’effort commun, équitablement réparti. En aucun cas cet effort ne doit pénaliser les communes vertueuses. tel mécanisme, nous préférons le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, tel qu’il est proposé par les rapporteurs, et dont les sommes ainsi mises en réserve seraient reversées aux collectivités contributrices. Par ailleurs, notre groupe ne souhaite pas qu’une part de péréquation soit conservée.

Enfin, nous accueillons positivement les évolutions apportées aux modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement, tout en estimant qu’une réforme globale reste nécessaire. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Indépendants votera les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, que s’est il donc passé depuis sept ans dans notre pays entre l’État et les collectivités territoriales ? Pourquoi tant de tensions inutiles ? Plus généralement, pourquoi, dans notre pays, est il aussi difficile d’avancer et de construire ensemble, alors que les grands défis auxquels l’État et les collectivités territoriales font face sont les mêmes ? Transition écologique, avenir de l’école, cohésion nationale, redressement des comptes publics, les sujets ne manquent pourtant pas. Les ministres des finances et du budget du précédent gouvernement n’ont eu de cesse de pointer du doigt la prétendue responsabilité des collectivités locales dans la dégradation des comptes publics. Tout le monde sait que c’était faux. Était ce pour détourner les regards de la mauvaise gestion budgétaire de l’État lui même, dont les déficits ont littéralement explosé depuis 2017 ? Probablement. soit, il n’y avait rien de tel pour braquer les élus locaux et rendre très difficile, voire impossible, tout partenariat avec l’État. En septembre dernier, une délégation de notre commission des finances s’est rendue au Japon. Quelle différence ! Et quelle surprise de constater que les relations financières entre l’État central et les collectivités locales n’y font l’objet d’aucune difficulté et sont régulièrement négociées dans des conditions à la fois sereines et constructives ! Je vous remercie donc, madame la ministre,

est la raison pour laquelle j’ai toujours dit que les collectivités locales devaient prendre une part à l’effort de redressement de nos comptes publics. Il ne serait du reste ni raisonnable ni responsable que seuls l’État et la sécurité sociale endossent les efforts nécessaires. Je salue le travail partenarial mené par notre commission des finances et le Gouvernement dans le cadre de ce budget. C’est exactement ce qu’il nous faut

est la raison pour laquelle le Sénat, sur l’initiative de notre commission des finances, a supprimé la disposition du PLF pour 2025 qui visait à réduire à la fois l’assiette et le taux du fonds de compensation pour la TVA. la raison pour laquelle notre commission des finances a proposé un dispositif de lissage conjoncturel des ressources des collectivités, désormais baptisé Dilico, qui nous semble plus pertinent, plus équilibré et qui sera certainement mieux accepté que le fonds de réserve proposé à l’article 64.

que, dans le domaine pourtant complexe des finances locales, nous gagnons tous à bâtir des dispositifs les plus lisibles possible, sans effet de seuil, fondés sur un faible nombre d’indicateurs et, surtout, reconnus et acceptés par tous.

Comme vous, je crois à l’État partenaire. Mais que doit on comprendre derrière la notion de partenariat, terme qui figure d’ailleurs dans l’intitulé de votre fonction ? Selon le,

qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation collègues : « tout en maintenant leur autonomie » ! Si nos collectivités ont bien entendu besoin d’autonomie, elles ont également besoin de stabilité et, surtout, d’un meilleur accompagnement.

Pour aider davantage les collectivités territoriales, je crois également que l’État et le Parlement doivent agir ensemble, afin de préserver un maximum d’investissements, avec un but clair : maintenir les emplois non délocalisables.

? Dans un esprit de compromis et de volonté de contribuer à l’apaisement des relations entre l’État et les collectivités, le groupe RDPI présentera enfin deux amendements.

Nous devons tous prendre notre part à l’effort national de réduction de nos déficits, mais cette part doit être juste et proportionnée aux moyens de chacune et de chacun. Dans la mesure où les collectivités subissent déjà de nombreuses contraintes financières, il nous faut trouver des solutions leur ménageant suffisamment d’oxygène.

? Enfin, notre pays sera t il un jour en mesure de permettre à chaque collectivité d’avoir les moyens de ses compétences ? Quoi qu’il en soit de ces éternelles interrogations, le groupe RDPI votera les crédits de cette mission, si nous en avons le temps. Je vous remercie,

Chaque année, qu’il s’agisse du projet de budget ou de nombreux autres textes, conformément à nos engagements et à notre ligne de conduite, nous rappelons et, surtout, nous prouvons, dans nos débats et dans nos votes, que le Sénat est le défenseur des territoires. En 2025, plus que jamais, ce rappel sera indispensable. La France est confrontée à un dérapage inquiétant de ses comptes publics, et des efforts sont nécessaires. Pas simplement pour complaire aux exigences des petits hommes gris des agences de notation, qui oublient de faire la leçon au Japon et aux ֤États Unis, lesquels connaissent respectivement une dette équivalente à 224 % et 120 % de leur PIB. Pas simplement pour corriger les excès d’un « quoi qu’il en coûte », que chacun de nous louait pourtant lorsqu’il s’agissait d’accompagner les ménages et les entreprises durant la crise de Pas simplement pour s’aligner sur les exigences de l’Union européenne, traduites en soustractions pour les collectivités et en additions pour les ménages. Vivre à crédit, être cigale, dépenser sans trop compter, c’est un euphorisant passager qui se transforme en poison pour les générations futures. Aussi, madame la ministre, le groupe RDSE se félicite de constater que le Gouvernement a entendu la voix de la sagesse, relayée par les heureuses paroles du président Larcher. Dans un premier temps, vous nous aviez présenté une facture indigeste obligeant les collectivités à procéder, sans discussion, à 5 milliards d’économies, alors qu’elles ne cessent de raboter leurs budgets pour pouvoir les voter en équilibre. Les dizaines de milliers de maires et les dizaines de milliers d’élus soumis à la fameuse règle d’or, qui leur interdit d’emprunter pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement, ont protesté. Leur colère, légitime, a t elle été réellement entendue ? La stabilité relative des enveloppes est en fait une diminution au regard de l’inflation, qui ne frappe pas seulement le panier de la ménagère. Car, faut il encore le répéter, nous demandons toujours plus et mieux aux communes, avec toujours moins.

Vous avez été élue locale, madame la ministre. Comment imaginer que le fonds instauré par l’article 64, rattaché à la mission des articles 30 et 31 du PLF qui enjoint à 450 collectivités de réaliser 14 milliards d’euros d’économies, serait sans effet sur les 35 000 communes françaises Associé au coup de rabot sur le reversement de fractions de la TVA, ce ruissellement à l’envers est un bien mauvais message adressé aux maires et aux élus, qui réalisent 70 % de l’investissement public dans notre pays

repousser la construction d’un giratoire, retarder la rénovation de l’éclairage public : la population trouvera là une nouvelle raison de dénigrer la déliquescence du service au public. Mais parce qu’ils sont dans l’obligation de voter des budgets en équilibre, que feront les élus pour entrer dans le carcan que vous imposez ? Supprimer la gratuité des cantines ? Augmenter les tarifs des transports publics ? Balayer les aménagements indispensables face au dérèglement et au changement climatiques, parce que vous réduisez le fonds vert comme peau de chagrin ? Les maires s’efforcent chaque jour, sous le feu croisé d’une multitude de normes et de contraintes, de trouver des solutions. Ils le font sans pleurnicher, sans gémir, sans quémander. fait de ce passif, et tout en regrettant que ce PLF fige des crispations et n’offre aucune perspective encourageante, au lieu de montrer un chemin d’espoir dans ce monde en décomposition, le RDSE décidera de son positionnement final après avoir parlementé.

Le Gouvernement avait fixé un objectif global de 40 milliards d’euros d’économies, dont 5 milliards d’euros à la charge des collectivités locales. Aussi, ce PLF a suscité de nombreuses interrogations du côté des collectivités territoriales. ont dû être entendues, car, oui, ce projet de loi est perfectible, comme l’a rappelé Michel Barnier à plusieurs reprises. Nous sommes ici pour cela ! Le PLF pour 2025 contenait trois mécanismes majeurs pour établir cette participation des collectivités à l’effort national. la création d’un fonds de réserve, à l’article 64. Ce mécanisme visait à prévoir un prélèvement sur les recettes fiscales des plus grandes collectivités. Le Sénat, par la voix de la commission des finances, a légitimement proposé de supprimer ce dispositif

Le reste de cette participation passait par deux dispositifs liés au FCTVA, examinés en première partie. À cet égard, le Sénat a été force de proposition en souhaitant Le contexte budgétaire contraignant oblige les collectivités à assumer une part équitable de l’effort national, mais une juste part. Les premières évolutions du Gouvernement sur ce sujet sont à saluer. Nous espérons continuer ce travail aujourd’hui et demain.

Dans ce cadre contraint, le maintien à un niveau élevé des principales dotations de soutien à l’investissement local est une mesure plus que bienvenue, qui ne réveille pas les vieux démons des années 2010.

Ce PLF pour 2025 reflète donc des arbitrages budgétaires complexes, mais nécessaires, pour l’avenir de notre pays, tout en préservant des dispositifs essentiels au soutien des collectivités territoriales. Aussi, le groupe Union Centriste votera les crédits de la présente présente mission. Madame la ministre, l’enjeu de l’année prochaine pour les collectivités réside dans une simplification des finances des collectivités, une refonte de la machinerie dantesque de la DGF et une meilleure lisibilité des ressources de chacun. Ce chantier est titanesque, nous le savons tous, mais nous appelons à le lancer au plus vite, pour que nous parvenions, en concertation avec les associations d’élus, le gouvernement en place et le Parlement, à trouver ce chemin de crête dont nos collectivités ont tant besoin. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » s’ouvre dans un contexte économique et budgétaire complètement inédit, sur fond d’instabilité politique majeure. Face à une dette colossale de 3 200 milliards d’euros, ce ne sont pas moins de 5 milliards d’euros de prélèvement sur les recettes des collectivités qui étaient initialement prévus. Si les collectivités locales sont prêtes à prendre leur part de l’effort national, cette décision a été particulièrement mal vécue par les élus locaux.

essentiel pour garantir l’avenir, une croissance économique durable et l’emploi local. Rappelons aussi que les collectivités appliquent scrupuleusement la règle d’or en votant des budgets à l’équilibre, en dépit d’une autonomie fiscale particulièrement mise à mal ces dernières années, avec des coupes budgétaires majeures, des suppressions de recettes très partiellement financées et des transferts de compétence qui n’ont fait que croître.

Pleinement consciente de ces aspects, je veux ici saluer le travail de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur général, qui a permis de rendre cet effort plus juste et proportionné en actant notamment la suppression de la réduction du taux du FCTVA, une mesure qui aurait touché de façon très inégale les collectivités. D’autres mécanismes, bien qu’ils contribuent à l’effort national, resteront lourds à porter. Le gel de la TVA affectée, qui se traduira par un effort de 1,2 milliard d’euros pour les collectivités, en est un exemple.

La rédaction proposée par le Gouvernement et l’architecture globale de ce dispositif posent de très nombreuses questions. Je souhaite que nos débats sur cette seconde partie du projet de budget nous permettent de trouver une solution plus juste et équitable, qui ne soit pas imposée aussi brutalement aux collectivités. Ce sera l’objet de l’un de mes amendements. Parallèlement, des ajustements demeurent nécessaires pour donner aux collectivités les moyens d’agir pleinement. À ce titre, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour attirer, une nouvelle fois, l’attention du Gouvernement sur l’absolue nécessité de revenir sur les modalités de recouvrement de la taxe d’aménagement. Avant 2022, cette taxe était exigible quelques mois après l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Mais depuis une réforme introduite dans la loi de finances pour 2021, c’est désormais la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qui est exigée pour déclencher le recouvrement de cette taxe.

L’article 61 du PLF modifie les modalités de détermination de la longueur de voirie prise en compte, à hauteur de 30 %, dans le calcul de la fraction « péréquation » de la DSR.

Retirer au législateur le pouvoir de déterminer la catégorie de voirie à retenir pour le calcul de la DSR, pour le renvoyer à un décret, remettrait en cause la légitimité même du critère de longueur de voirie ! Ce serait particulièrement préjudiciable aux communes rurales, pour lesquelles l’entretien de la voirie est très coûteux. Nous défendrons donc un amendement tendant à supprimer cette mesure injuste. J’en viens Si les collectivités doivent participer au redressement des comptes publics, notre groupe considère qu’il faut que cette contribution repose sur un principe intangible de justice territoriale. C’est pourquoi nous approuvons la proposition de la commission de fonder le prélèvement sur des critères objectifs de richesse des territoires, ainsi que le glissement sur trois ans du reversement et sa réduction à 1 milliard d’euros. C’est aussi ce principe de justice territoriale qui nous a amenés à voter, en première partie, la suppression de la baisse prévue de 10 % du FCTVA et le maintien du périmètre d’éligibilité cette mesure percuterait directement l’investissement porté par les collectivités, alors qu’il est essentiel au maintien du tissu économique et social dans tous les territoires de France.

Cette disposition serait à haut risque pour les communes rurales, dont la recette du foncier non bâti représente parfois plus de la moitié de la recette fiscale totale de la commune.

Je souhaite revenir quelques instants sur le sujet de la DGF. Nous approuvons l’augmentation de la péréquation à hauteur de 320 millions d’euros que propose le Gouvernement. En revanche, accroître la péréquation à enveloppe constante

ci a été utilement réformée en 2024 – cela a été rappelé. Toutefois, l’élargissement des critères d’éligibilité a conduit à maintenir des niveaux de dotation très peu élevés dans de nombreuses communes. C’est pourquoi nous proposons sa revalorisation à hauteur de 10 millions d’euros. Nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur tous ces sujets au cours de nos débats, avec l’objectif, pour ce qui nous concerne, de voter les crédits de la mission. La parole

ne suis pas le premier à le rappeler ! Dans ce contexte difficile, il est impératif de rappeler le rôle essentiel des collectivités, qui sont dans leur ensemble garantes des services publics de proximité et acteurs incontournables de l’investissement public. Le Sénat s’est engagé, lors de l’examen de ce projet de budget, à en modifier le contenu en faveur d’une participation plus juste et proportionnée des collectivités à l’effort budgétaire. Concrètement, le PLF pour 2025 maintient globalement la stabilité des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », ce qui traduit la volonté du Gouvernement de soutenir l’investissement local.

le verdissement des dotations d’investissement, avec l’augmentation des crédits pour les projets environnementaux, je constate que les gouvernements successifs ne tiennent pas suffisamment compte du risque d’un fléchage excessif des dotations, qui réduit les marges de manœuvre des collectivités. Ce fléchage doit être réaliste et incitatif, comme nous l’avons décidé, par exemple, à propos du fonds vert, à la condition qu’il reste à la main des préfets. S’agissant des départements, le Gouvernement propose des mesures pour atténuer l’effort budgétaire qui leur est demandé Ces mesures, bienvenues, ne doivent pas masquer les difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les départements, notamment en matière de dépenses sociales – je pense au secteur du grand âge.

Les communes rurales, confrontées à des défis spécifiques, doivent bénéficier d’un soutien accru. L’ingénierie en milieu rural mérite une attention particulière pour permettre aux communes de monter des projets et d’accéder aux financements. De même, les lignes d’aménagement du territoire territoire doivent être écartées de l’éventuelle mise en place d’une taxe de solidarité sur les billets d’avion, pour des raisons évidentes de continuité territoriale. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, j’avais insisté sur l’affaiblissement des marges de manœuvre fiscales des collectivités et la fragilisation de leur autonomie financière. Le contexte actuel renforce ce constat. Il impose de mettre en œuvre une refonte des relations entre l’État et les collectivités territoriales, fondées sur la confiance, la responsabilité et la différenciation. En ce sens, je crois pouvoir

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur

Ce dispositif a permis de compléter ce que le gouvernement de Michel Barnier avait proposé pour conjuguer les spécificités des collectivités territoriales avec la nécessité du redressement des finances publiques. parvenus au terme de nos discussions, je note que les conditions de préparation du budget – la dernière ligne droite de notre dialogue – n’ont probablement pas permis au Gouvernement de trouver, en ces derniers moments de débat, un accord final avec le Sénat.

reversés aux collectivités ayant contribué. Monsieur Chevalier, nous ne parlons donc plus de péréquation, et, bien évidemment, les communes d’outre mer éligibles seront toutes exonérées. Quel que soit le système que choisira votre assemblée, il devra être être lisible et juste. Surtout, il lui faudra apporter la garantie d’une participation réelle des collectivités territoriales à la réduction du déficit.

que les crédits ouverts au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » soient stables. Cette stabilité est le signe que l’État continue d’accompagner les collectivités

qu’il s’agisse des zones rurales, des quartiers relevant de la politique de la ville ou des territoires ultramarins et insulaires. Cet accompagnement vise à renforcer leur capacité à porter des projets structurants

entre l’État et les collectivités. Notre deuxième objectif est de garantir des ressources pérennes et adaptées aux collectivités territoriales en cas d’événements imprévus, notamment par leur ampleur,

l’exercice 2025 permettra d’accompagner le financement des travaux. Notre troisième objectif est de compenser les charges transférées aux collectivités dans le cadre de la décentralisation,

(DSU) bénéficie d’une majoration de 140 millions d’euros, tandis que la dotation de solidarité rurale augmente de 150 millions d’euros.

Élue parmi les élus, je mesure évidemment la complémentarité de chaque strate, la spécificité et la singularité de chaque territoire, qu’il soit rural, urbain, hexagonal, insulaire ou ultramarin. Mesdames, messieurs

Mes chers collègues, je vous rappelle que, pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximale de la discussion à huit

de collectivité – bloc communal, département et région –, en fonction du poids des recettes réelles de fonctionnement et de l’épargne brute. Les communes contribueraient ainsi à hauteur de 255 millions d’euros, de même que les EPCI ; les départements,

Les communes et EPCI contributeurs seraient définis en fonction d’un indice synthétique composé de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant. Seules les communes et EPCI dont l’indice est supérieur à 110 % de la moyenne nationale La contribution serait répartie de manière très progressive entre les communes contributrices, de telle sorte qu’aucun effet de seuil ne subsiste. Les communes exonérées du Fonds national de péréquation des ou à la DSU seraient exonérées. De même, afin d’éviter des contributions négligeables, les communes dont la contribution serait inférieure à 1 000 euros ne seraient pas soumises au dispositif. En ce qui concerne les départements, seuls ceux

aucun effet de seuil n’existant entre le dernier département exonéré et le premier département contributeur. Enfin, la contribution des régions serait répartie selon la contribution au titre du fonds de solidarité régionale. Les régions d’outre mer et la Corse en seraient exonérées. Les contributions seraient reversées aux collectivités contributives pendant trois ans, à raison d’un tiers par an. Il s’agit donc d’une mise en réserve, et non d’une ponction. Les simulations dont nous disposons – nous les avons élaborées avec les services de la ministre, que je remercie

par l’Observatoire des inégalités. Nos communes et nos EPCI, qui participent aux politiques publiques et qui sont les portes d’entrée des demandes de nos compatriotes, sont injustement mises à contribution.

parties prenantes, comme les Français et comme les entreprises, à l’effort de redressement des comptes publics. Or je souhaite en cet instant rappeler les propos

Merci,

», mes chers collègues – il faut être réaliste et, une fois n’est pas coutume, un peu politique. Je ne sais pas ce qu’il se passera dans deux heures. Je ne sais pas qui sera au Gouvernement demain. Je ne sais pas

Le scrutin est clos.

Le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT), actuellement fixé à 187 millions d’euros, ne suffit plus à couvrir les coûts croissants de cette continuité. Des soutiens exceptionnels de 33 millions et de 40 millions d’euros ont été accordés en 2022 et 2023 au travers des précédentes lois de finances.

constitue une dotation spécifique, qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité et à garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’île et le continent, notamment en matière de transport aérien et maritime.

Je connais, madame la ministre, votre attachement à la Corse. Alors que le montant demandé est inférieur à la perte de recettes causée par la non réévaluation de la

intercommunales et communales – pour assurer une allocation en fonction de critères de ressources et de charges. Les collectivités disposent donc toujours de la possibilité d’orienter ces ressources libres d’emploi vers les politiques publiques de leur choix. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

des départements –, soit près de 2 milliards. Cet amendement vise à minorer ces ouvertures de 55 millions d’euros pour tenir l’objectif du Gouvernement de ramener le déficit à 5 % du PIB en 2025. Cette minoration n’aura pas d’effet sur le montant effectivement disponible en 2025 pour le soutien des projets des collectivités. Très concrètement, comme le Gouvernement l’a expliqué préalablement, cette annulation sera portée pour moitié par la DSIL et pour moitié par la DETR. Elle n’entraînera donc pas de réduction des autorisations d’engagement mises à la disposition des préfets en 2025 pour soutenir les projets d’investissement des collectivités. La réserve de précaution habituellement portée par ces dotations, décidée en début d’année budgétaire et qui fait l’objet d’une annulation partielle ou totale en fin d’année, sera réduite

Comme chacun le sait, la DETR est une dotation essentielle au financement des projets d’équipement public dans les zones rurales, comme la construction d’infrastructures ou la rénovation de bâtiments publics. publics. Elle joue un rôle stratégique dans la réduction des inégalités territoriales en permettant aux communes rurales de bénéficier d’un soutien financier équitable pour des projets essentiels à leur développement. Cet amendement vise à revaloriser la DETR en 2025, afin de l’adapter à l’évolution prévisionnelle de l’inflation, soit une augmentation de 1,8 %. Un tel dispositif permettrait de compenser la hausse des coûts de construction et de préserver la capacité des collectivités locales à financer leurs projets. Cette revalorisation viendrait également répondre aux préoccupations des élus locaux, qui dénoncent régulièrement une érosion du pouvoir d’achat lié aux dotations face à une inflation persistante. Quel est l’avis de la commission ? Compte tenu

la réalisation de ces plans est parfois complexe : « Les élus de communes rurales ont également alerté la mission d’information sur le manque de ressources humaines comme techniques à l’échelle de la commune pour la réalisation du plan communal de sauvegarde, obligeant certaines communes à déléguer ces missions à des prestataires externes. Beaucoup d’élus locaux souhaiteraient ainsi pouvoir bénéficier d’un accompagnement plus poussé de l’État en matière d’ingénierie, afin de pouvoir être plus à même de développer ces outils par eux mêmes. De même, les exercices anti incendie représentent un coût difficilement pris en charge par les collectivités, alors que leur utilité dans la lutte contre les feux de forêt est avérée. C’est pourquoi cette mission d’information recommandait d’inclure dans la dotation d’équipement des territoires ruraux une ligne budgétaire spécifique au financement des plans communaux de sauvegarde. Si la plupart des départements mettent en avant un taux de couverture autour de 75 % ou de 80 %, de nombreuses communes, souvent les plus petites, qui disposent de moins de moyens, sont encore dépourvues de plans communaux de sauvegarde (PCS), et ce en dépit de la multiplication et de l’intensification des catastrophes naturelles. À cela s’ajoute le fait que de nombreuses communes n’ont pas de PCS, car il n’y a pas de risque identifié sur leur périmètre. Or, le changement climatique faisant émerger des vulnérabilités nouvelles, il est important que toutes les communes en soient dotées. Il me semble important d’envisager de les accompagner dans ce sens.

Augmenter le montant de la dotation d’équipement des territoires ruraux de 10 millions d’euros pour permettre le financement des plans communaux de sauvegarde en diminuant un programme d’investissement

le projet de loi de finances pour 2024. La nouvelle dotation, abondée à hauteur de 100 millions d’euros, est destinée à toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. Ce dispositif s’inscrit dans un mouvement vertueux de reconnaissance du rôle joué par les communes

de préservation de la biodiversité ou de lutte contre le réchauffement climatique. En 2019, une première étape a été franchie avec la création d’une dotation commune appelée dotation de soutien aux

de la protection de l’environnement. Or la préservation de ces espaces naturels – ô combien importants, madame la ministre, vous le savez, puisque votre gouvernement a inscrit ses pas dans ceux de ses prédécesseurs pour augmenter la part du territoire national protégé – réclame

Le nombre de bénéficiaires est passé, lui, de 6 388 communes en 2023 à 8 921 communes, comme l’a rappelé votre rapporteur. Les crédits de l’action du programme 122, qui ont vocation à aider les collectivités territoriales confrontées à des circonstances exceptionnelles, ne sauraient être utilisés pour financer une augmentation du montant de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Par ailleurs, la pérennisation de cette dotation à hauteur de 100 millions en 2025 et l’élargissement du périmètre des espaces protégés retenus représentent déjà un effort considérable de l’État dans le contexte aujourd’hui dégradé des finances publiques. Au regard de ces éléments, le Gouvernement

les périmètres de protection de captages d’eau A qui sont l’objet de contraintes environnementales extrêmement fortes. Il paraît souhaitable que les communes qui les subissent puissent obtenir des compensations au travers de cette dotation.

dans l’actuel contexte dégradé des finances publiques : avis défavorable.

les présidents des deux associations de maires de Nouvelle Calédonie. Mes chers collègues, les besoins des communes sont énormes. On les chiffre à plus de 180 millions d’euros : 64 millions d’euros pour la reconstruction, 54 millions de pertes sur le fonctionnement des communes, 13 millions d’euros de baisses liées à la perte d’autres recettes de fonctionnement, 50 millions de pertes sur la fiscalité additionnelle. En Nouvelle Calédonie, ce bout de France, ce caillou, il y a aujourd’hui des gens qui sont en train de manquer de nourriture.

Il s’agit de renforcer les capacités d’action de la collectivité, qui sont essentielles au soutien socio économique du territoire martiniquais. En 2023, la CTM a soutenu 1 300 entreprises, 50 associations sportives, 120 associations culturelles et a fourni des prestations à des milliers de bénéficiaires. La période actuelle est marquée par un contexte de crise, lié à la vie chère, à une précarité accrue et au retrait de certaines interventions de la CTM, premier partenaire de l’État au plan local, qui assure à la fois les compétences d’une région et d’un département. La CTM envisage, par ailleurs, un plan de restructuration, avec la révision d’un certain nombre de ses guichets et une revue de ses dépenses de fonctionnement et, par la suite, des actions de réduction importantes – immobilier, personnel, achats, etc. Ces restrictions affecteront inévitablement le service public et limiteront l’investissement public local sur l’île, dont la CTM assure les deux tiers. Toutefois, le souhait des élus de la CTM est de maintenir le soutien aux personnes vulnérables et un niveau d’investissement qui garantisse la prise en compte des priorités pour l’avenir du territoire, notamment l’urgence de la sécurisation des collèges et des lycées, avec une programmation pluriannuelle d’investissement fixée à 200 millions d’euros par an, ainsi que le lancement d’un budget vert. Ces objectifs demeurent conditionnés à la capacité de financement autonome de la CTM, laquelle reste insuffisante en l’absence de soutien de l’État. Cet amendement vise à octroyer une dotation d’amorçage en fonctionnement de 50 millions d’euros pour compenser l’absence de soutien initial de l’État et aider la CTM à répondre aux besoins structurels et socio économiques urgents de la Martinique. Cet amendement a été élaboré avec la collectivité territoriale et l’Association des régions de France.

au profit des collectivités qui ont été intégrées dans le périmètre des variables d’ajustement pour gager, au sein de l’enveloppe normée, la hausse de certains concours financiers par la baisse corrélative des autres. Pour chaque taxe, nous pouvons donc différencier des dispositifs d’exonération. Le montant exonéré correspond à la perte de recettes avant compensation par l’État pour les collectivités liée à la mise en œuvre d’un dispositif d’exonération de droit.

Le coefficient de minoration amalgamé est appliqué au montant de l’allocation avant minoration pour obtenir le montant de l’allocation versée par l’État aux collectivités. Il s’est élevé à 43 millions d’euros pour les communes en 2023. Deuxièmement, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) font l’objet d’une compensation par l’État ajustée aux nécessités de la rigueur budgétaire. Vous le savez, cette compensation est égale au produit des bases exonérées l’année précédente par le taux de TFPB en vigueur l’année précédente. Le produit est minoré par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’en 2017 en loi de finances. Selon le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux remis en 2024

Par ailleurs, le Gouvernement est allé au devant de la compensation des seules pertes de recettes induites par des allégements fisco additionnels, en aidant les communes et les EPCI qui subissent une perte soudaine de TFPB par l’article 138 de la loi du 29 décembre 2023, qui a souhaité couvrir par une compensation spéciale dégressive les communes et EPCI à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de bases de TFPB liée à la délocalisation de locaux industriels et à la volatilité de leurs bases. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable

En 2020, un fonds de péréquation a été mis en place. Son montant est estimé à 1,4 milliard pour 2025, contre 1,9 milliard d’euros en 2024, soit 500 millions de moins. De nombreux départements seront en difficulté. En 2024, un fonds de sauvegarde

Mes collègues ont raison de rappeler la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les départements aujourd’hui. Je crois que l’on ne peut que souscrire à leurs propos. Néanmoins, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements,

Merci,

M. Guy Benarroche. Le programme 122 regroupe les aides spécifiques aux collectivités, avec comme objectif de garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation de ces dernières en cas de catastrophe naturelle. Les autorisations d’engagement de ce programme sont aujourd’hui

loi de finances prévoit une diminution des crédits en faveur des subventions pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques et que l’ensemble des crédits ouverts à la suite de la tempête en Bretagne sont désormais consommés, la solidarité nationale doit de nouveau fonctionner pour les territoires qui ont subi de nouvelles intempéries ces derniers mois.

s’élever à plus de 60 millions d’euros. Grâce aux services de secours et à la préfecture, le pire a pu être évité, mais il est désormais temps de reconstruire et, surtout, de reconstruire autrement pour éviter que des dégradations du même ordre n’adviennent Pour cela, les collectivités territoriales, qui ont assisté depuis plus de sept ans à une baisse continue de leurs dotations, doivent être soutenues dans les meilleurs délais. Ces démarches s’inscrivent pleinement dans le plan national d’adaptation au changement climatique, qui a été présenté ici par le Gouvernement à la fin du mois d’octobre. D’ailleurs, une délibération sera présentée demain au conseil métropolitain de Saint Étienne Métropole pour demander la création d’un fonds d’aide exceptionnel en faveur des communes reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite des événements climatiques du mois d’octobre. Madame la ministre, les collectivités sont prêtes à agir pour une reconstruction ambitieuse. L’État doit être à leurs côtés ! L’amendement

afin de mieux répondre à la recrudescence des violences, menaces et outrages auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. Aujourd’hui, la protection fonctionnelle ne s’applique qu’aux membres des exécutifs, à l’exclusion de tous les autres élus, ce qui constitue une inégalité de traitement. Le Sénat Le Sénat s’est lui même saisi de cette situation, puisqu’il a intégré, dans sa proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, adoptée en mars dernier, une disposition ouvrant le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus, sous conditions.

Comme vous le savez, la réponse à ce problème dépasse largement le cadre budgétaire. Nous sommes appelés à consolider l’arsenal répressif en cas de violences commises à l’égard

élu local » (DPEL) a été abondée de 22 millions d’euros en deux ans. La loi de finances pour 2024 a étendu, la DPEL, la prise en charge de la protection des élus pour l’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants. Un plan de lutte contre les violences faites aux élus a été doté de 5 millions d’euros Le financement d’une nouvelle mesure de 50 millions d’euros n’est pas soutenable, surtout si elle est financée par une minoration des crédits du programme 119, qui relève de dotations constitutionnellement dues aux collectivités. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable

pour le développement d’activités périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Il permet un cofinancement entre l’État et les collectivités pour les temps d’animation. Selon France Urbaine, entre 2022 et 2023, 1 262 communes en ont bénéficié, pour un total de 41 millions d’euros. La suppression de ce fonds, annoncée en 2024 et programmée par le Gouvernement, mettrait en péril l’équilibre financier des communes et leurs politiques d’éducation et d’inclusion à destination des enfants et de l’ensemble des habitants. Cet amendement vise à soutenir les collectivités, les acteurs de l’animation périscolaire et les familles

dans la fonction publique territoriale, précisée par décret en 2024, introduit une obligation, pour les employeurs territoriaux, de contribuer aux couvertures santé et prévoyance de leurs agents. Pour la collectivité employeuse, le coût sera acquitté en deux fois : en 2025 et en 2026. Il sera de 22 euros par agent

spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) les contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique d’État ou territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. souci de parallélisme avec ce qui se fait dans le privé. Ce dispositif a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement. Certes, il ne couvre pas l’ensemble du coût de la prise en charge de la protection sociale complémentaire, mais dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons, ce compromis me semble acceptable. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements. Quel

sont victimes d’insultes, de menaces et, souvent, d’agressions physiques. Face à cette situation,

Pour mémoire, l’article 21 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoyait de ne plus soumettre à la taxe communale sur les spectacles les droits d’entrée perçus par les organisateurs de manifestations sportives. En parallèle, un prélèvement sur recettes de l’État avait été institué pour compenser les pertes subies par les communes, d’un montant égal au produit perçu au titre de l’année 2013. Ce dispositif ne tenait cependant pas compte de la situation des communes qui, bien que ne percevant pas la taxe sur les spectacles au titre des manifestations sportives en 2013, et qui n’étaient donc pas éligibles au prélèvement sur recettes (PSR) de compensation, s’étaient engagées dans des projets d’investissement en équipements sportifs de grande ampleur. Or elles comptaient précisément sur ces recettes pour assumer la charge financière de tels équipements. Cet amendement tend donc à combler cette lacune du dispositif initial en instituant une dotation

rectifié. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », figurant à l’état B. Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

ces crédits, modifiés. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. Par lettre en date du 6 novembre, M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’espace réservé à son groupe du jeudi 19 décembre de la proposition de résolution, en application de l’article 34 1 de la Constitution, appelant à l’introduction de la proportionnelle pour les élections législatives. Acte est donné de cette demande. Pour l’examen de cette proposition de résolution, les interventions des orateurs vaudront explications de vote.

n° II 68 rectifié. Cet amendement concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population en dessous de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur part de DGF en raison de la perte d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine. Il tend à renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées en lissant les pertes subies sur une période plus longue

Mme Sylviane Noël. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les communes représentant 15 % de la population du canton reçoivent la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent plus en bénéficier.

lorsque la commune chef lieu de canton de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1 janvier 2014. L’amendement

semble comporter une lacune, dans la mesure où sa rédaction ne permet pas d’assurer que, avant la fusion, le chef lieu comptait moins de 10 000 habitants. Par ailleurs, la commission est attentive à la simplicité et à l’intelligibilité de la norme.

du Gouvernement ? La fraction bourg centre de la dotation de solidarité rurale est destinée, par des attributions importantes, à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural. Les critères qui lui sont

collectivités communales plus fortes et plus dynamiques, en mesure d’exercer davantage de compétences et de supporter plus de charges. Il n’y a donc pas de raison pour que ce dépassement du seuil de population par une commune nouvelle

si au moins l’une de ses communes fondatrices bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2023, cette mesure exceptionnelle ne concernait que deux communes nouvelles, qui avaient perdu des montants très significatifs de DGF.

C’est pourquoi, afin de compléter le pacte de stabilité de la DGF de ces communes nouvelles, qui représentent des cas très particuliers – seules deux sont concernées –, le présent amendement vise à maintenir le montant

Or une commune nouvelle n’est pas éternellement nouvelle ; après plusieurs années, elle redevient une commune comme les autres… En outre, la loi de finances pour 2024 a créé une dotation spécifique pour les communes nouvelles, comme vous l’avez rappelé, financée par un prélèvement sur les recettes de l’État.

de 34 % à la moyenne nationale. La loi de finances pour 2024 a institué une dotation en faveur des communes nouvelles, distincte de la DGF, qui permet déjà de compenser toute perte pour les communes nouvelle à la suite d’une fusion. Un nouveau mécanisme de garantie au sein de la DGF ne nous paraît pas utile

en passant sous le seuil des 10 000 habitants et qui ne l’a pas retrouvée en 2023 lorsque sa population a de nouveau dépassé les 10 000 habitants. Pour autant, cette commune a bénéficié d’une hausse de 4 % de sa DGF en 2024, du fait d’une augmentation de 15 % de sa dotation nationale

Il vise à adapter le calendrier d’application des nouvelles modalités de calcul de l’effort fiscal, redéfinies en 2022 à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Le nouveau mode de calcul devait initialement entrer en vigueur dès 2023, selon un calendrier progressif. Cependant, en supprimant du calcul de l’effort fiscal la prise en compte des produits fiscaux intercommunaux, la définition retenue en 2022 induit des effets de biais non satisfaisants, pénalisant en particulier les communes membres d’EPCI plus fortement intégrés. Le PLF pour 2025 ne comporte aucune disposition spécifique sur ce sujet ; par conséquent, l’application du nouveau mode de calcul devrait être portée à 40 % l’an prochain, conformément au rythme prévu initialement. Ce passage de 10 % en 2024 à 40 % en 2025 représenterait une marche élevée, produisant des effets négatifs importants sur les dotations des communes les plus pénalisées par la nouvelle définition. De telles incidences négatives seront particulièrement malvenues en ce qu’elles s’ajouteront aux conséquences du gel de la DGF en 2025.

n° II 47 rectifié. Le présent amendement vise à mettre fin à une doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle

effort ! Il vise à prévoir que le financement de la péréquation verticale sera assuré par les communes à haut potentiel financier. La commission des finances n’est pas favorable à ce dispositif qui aurait pour conséquence d’accroître les prélèvements des collectivités

Les habitants des communes rurales sont donc bien, et de très loin, les principaux bénéficiaires de la DETR. L’adoption de cet amendement conduirait à rendre inéligibles à cette dotation 3 320 communes, soit 10 % des communes actuellement éligibles, dont 2 000 communes de moins de 5 000 habitants, où les services publics bénéficient à des populations rurales.

certaines communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire, en dépit des

Le Gouvernement souhaite donc abroger cette interdiction de cumul en actant le principe selon lequel, sous réserve des règles de participation minimale du maître d’ouvrage, les dotations d’investissement, dont la DETR, sont bien toutes cumulables entre elles.

pour présenter l’amendement n° II 350 rectifié. Les maires, particulièrement dans les petites communes, croulent sous les contraintes bureaucratiques. Pour une simple demande de DETR, il faut parfois constituer des dossiers de plusieurs dizaines de pages, rassembler une multitude de pièces justificatives, dont certaines sont redondantes ou d’une utilité discutable.

cet amendement, il est proposé deux leviers d’action pragmatiques. Tout d’abord, nous souhaitons confier à la commission d’attribution de la DETR un nouveau rôle de proposition en matière de simplification. Qui mieux que cette instance, qui examine plusieurs centaines de dossiers chaque année, peut identifier les complexités inutiles et suggérer des pistes d’amélioration Ensuite, nous demandons au Gouvernement de produire, d’ici à septembre 2025, une évaluation complète des contraintes actuelles et de proposer des mesures concrètes d’allégement. Il s’agit non pas de supprimer tout contrôle, mais simplement de rendre les procédures plus efficaces. Chaque heure que les secrétaires de mairie passent à constituer des dossiers administratifs

l’amendement n° II 369. Les commissions d’élus de la DETR présentes dans chaque département ne consultent les élus que sur les subventions dont le montant dépasse 100 000 euros. Dans un souci de renforcer l’implication des élus dans les décisions de l’État et de ses représentants concernant l’attribution de la DETR, cet amendement vise à abaisser ce seuil à 50 000 euros.

pour que les élus puissent participer activement à la défense de leurs projets. Bravo

les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour les déposer. Afin de leur permettre de constituer leur dossier dans de meilleures conditions, cet amendement vise à faire disposer les communes d’un délai minimal à compter du lancement des appels à projets départementaux.

des subventions au second semestre alors qu’ils devaient auparavant notifier l’intégralité des subventions avant la fin du premier semestre. L’idée était de retrouver un peu de souplesse, de manière à financer des projets déposés tout

Mme Sylviane Noël. Nous constatons dans nombre de départements une évolution des pratiques administratives : celles ci imposent désormais aux collectivités locales d’atteindre le stade de l’avant projet pour pouvoir déposer une demande de subvention, ce qui constitue une entrave importante pour les collectivités locales.

Outre les difficultés à monter les dossiers, le suivi des demandes pose aussi des problèmes au sein de nos collectivités. Alors que les marges de manœuvre financières des communes tendent à se resserrer, les maires ont de plus en plus besoin de visibilité et doivent avoir la certitude de disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets.

et de territorialisation de la transition écologique. Ces dispositions n’instaurent pas un mécanisme d’écoconditionnalité dans l’attribution des subventions ; elles visent seulement à inciter les collectivités et à encourager les projets vertueux pour l’environnement, pour un montant total de 520 millions d’euros sur près de 2 milliards d’euros de dotations d’investissement. Comme je le disais tout à l’heure, la DSIL est une dotation polyvalente, qui vise à soutenir de nombreuses politiques publiques locales. Le Gouvernement souhaite donc qu’un projet d’investissement puisse être soutenu même s’il ne contribue pas directement à la transition